d’observation ?… Le procès verbal est adopté sous les réserves d’usage. L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote à la tribune du projet de loi de finances pour 2024,

plus tard. L’inflation parlementaire, de 175 %, dépasse très largement l’inflation monétaire ! Il est grand temps que notre autorité de régulation mette fin à cette politique expansionniste. Nous n’avons malheureusement plus de marges de manœuvre.

et commencer à rembourser notre dette, dont la charge d’intérêt explose. L’achoppement des discussions du conseil Écofin sur la révision du pacte de stabilité et de tout particulièrement sur les modalités du bras correctif, soit les efforts demandés aux États membres en procédure de déficit excessif, montre combien la position de la France est fragilisée sur la scène européenne du seul fait de ses mauvais résultats économiques. La majorité sénatoriale a fait de la politique, dans le bon sens du terme. Nous avons été capables de proposer des choix responsables, « à l’euro près

il s’agit bien d’un accompagnement vers la fin de la politique du chèque. Il faudra cependant penser à une réforme, car une partie de la population ne pourra pas payer de manière durable de l’électricité à plus de 220 euros par mégawattheure. Nous avons également refusé la création d’un paradis fiscal pour la Fifa.

ne se feront pas au détriment du défi de la transition écologique ou de la croissance. Ce sont de vraies économies, pas des économies de papier. L’effort de redressement des finances de l’État est réel, et non porté exclusivement par la disparition progressive et inéluctable des mesures de crise. Cet effort permet d’avoir un déficit public inférieur à 3 % dès 2025. Notre trajectoire pour la loi de programmation des finances publiques est réaliste,

Le Sénat a voté des dispositions vous permettant de mettre en œuvre ce « pari de la confiance », ce pari de la réussite de l’action décentralisée. Permettez moi le fonds climat territorial, l’affectation d’une fraction du produit des quotas carbone aux autorités organisatrices de la mobilité, le maintien du prêt à taux zéro (PTZ) dans le neuf sur l’ensemble du territoire, une meilleure définition des (FFR). Avant de voter en faveur de ce projet de loi de finances, le groupe Les Républicains a quelques regrets, qui ont notamment été exprimés lors des explications de vote de la première partie. Je pense notamment au rejet de la hausse du plafond

vous propose d’ores et déjà quelques sujets : la taxe de séjour, la fiscalité de la location de courte durée, les ressources des chambres consulaires, la réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, la réforme de la fiscalité de l’eau. La condition du succès est le partage de l’information. Quand aurons nous connaissance des fiches d’évaluation des dépenses fiscales arrivées à échéance ? Monsieur le ministre, vous trouverez encore face à vous, l’année prochaine, une opposition attentive, mais constructive sur les travées du groupe Les Républicains, pour rendre possible ce qui est nécessaire, pour une France tournée vers l’avenir.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le dernier budget de l’État en excédent a été voté fin 1973. C’était il y a cinquante ans, sous Georges Pompidou. Après les Trente Glorieuses, nous bouclons les « Cinquante Piteuses », avec un déficit de 144 milliards d’euros pour l’année à venir. François Fillon, alors Premier ministre, avouait en 2011 qu’il était « à la tête d’un État en faillite ». Il y avait alors 1 500 milliards de dettes. Que devrions nous dire de notre situation actuelle, la dette ayant plus que doublé pour atteindre les 3 000 milliards ? La seule charge de la dette explosera à 52 milliards d’euros l’an prochain. Elle risque de devenir le premier poste budgétaire, devant l’éducation nationale. Notre endettement représentera près de 110 % du PIB en 2024, alors qu’il était de 98 % en 2017. Depuis 1973, à défaut de poches de pétrole en France, les gouvernements successifs ont décidé de faire les poches des Français. Et le forage fonctionne à plein régime. Aujourd’hui, les prélèvements obligatoires en France représentent 48 % du PIB ! Sur 100 euros de production de richesse, 48 euros vont à la sphère publique. C’est 6,3 points de plus que le taux moyen des autres pays européens. Au vu de ce record, vos marges de manœuvre sont nulles. Vous ne parviendrez pas à désendetter le pays, lutter contre l’inflation et investir pour l’avenir sans remettre en question le système économique actuel de socialisme tentaculaire à l’intérieur du pays … Si seulement ! … et de libéralisme sans entrave à l’extérieur ! Pour retrouver de la croissance, il faut moins d’impôts et de normes pour développer nos industries, réduites de moitié depuis les années 1970, et moins d’accords de libre échange, comme celui entre l’Union européenne et le Mercosur, en cours de négociation,

votre gouvernement, qui survit grâce à sa perfusion permanente de 49.3, a daigné supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et pour cause ! Cette baisse d’impôts viendra grever non pas son train de vie, mais le budget des collectivités territoriales, déjà exsangue. C’est tout bonnement irresponsable Il n’y a plus d’État stratège, plus d’investissement stratégique, malgré un haut commissariat au plan, pas de réindustrialisation viable, pas de plan d’infrastructures. L’État doit se réformer pour parvenir à un libéralisme national : libérer à l’intérieur et protéger à l’extérieur. Emmanuel Macron avait promis « 60 milliards d’économies par an » en 2017 ; il a aggravé la dette de 700 milliards d’euros. Édouard Philippe a parlé d’« addiction française à la dépense et nous avons eu le « quoi qu’il en coûte » macronien, pour que, le ministre de l’économie finisse par planter le dernier clou dans le cercueil du mythe du Mozart de la finance, en avouant que nous sommes finalement « à l’euro près ». Il faut conclure, mon cher collègue. En tant que sénateur, dont la fonction est celle de contrôler ce que vous faites de l’argent du contribuable, je m’opposerai bien évidemment à ce projet de loi de finances pour 2024. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

ce dimanche, Javier Milei est officiellement devenu le nouveau président de la République argentine. C’est la première fois qu’un candidat autoproclamé « libertarien » arrive aux plus hautes responsabilités. Le populisme et le dégagisme ont trouvé un nouveau carburant : la réduction radicale des dépenses publiques. Une image a marqué la campagne de Milei. On le voit rugir comme un fou en brandissant une tronçonneuse. Le nouveau président promet de juguler l’inflation en tronçonnant la dépense publique. Le message est on ne peut plus clair : « Ça va saigner Dans la première qu’il a donnée après son élection, Milei a déclaré : « L’équilibre budgétaire est non négociable. C’est zéro déficit. Si un ministre présente un budget en déficit, je le vire. » Je veux rassurer tous mes collègues qui redoutent sans cesse « l’Internationale de l’ultralibéralisme ». La France en est encore loin ! Il faudrait d’abord qu’elle se réconcilie avec le libéralisme. Le projet de loi de finances pour 2024 n’a rien d’un budget à la tronçonneuse ; c’est le moins que l’on puisse dire. C’est un budget pragmatique, qui nous ramène lentement, mais sûrement dans les clous de nos engagements européens. Les dépenses ont augmenté, la dette aussi, mais le déficit est contenu en deçà de 4,5 %, et l’inflation est limitée à 2,6 %. On est loin de l’austérité qui s’annonce sous les cieux argentins. Le texte du Gouvernement place la France sur une trajectoire raisonnable, qui nous laisse encore espérer un retour à la normale sans ajustement brutal. La commission des finances a proposé d’accélérer un peu le rythme. Monsieur le ministre, si vous choisissiez de suivre le train sénatorial, vous arriveriez un peu plus vite à votre objectif de maîtrise des dépenses publiques. vous avons fait de nombreuses propositions pour limiter la hausse des dépenses. C’est le cas sur la mission « Travail et emploi », dont j’ai l’honneur de rapporter les crédits avec ma collègue Ghislaine Senée. Le recentrage de l’apprentissage sur les artisans et les PME permettrait de réaliser 725 millions d’euros d’économies par an. Cela mérite que l’on s’y intéresse.

Je serai très clair : l’essor de l’apprentissage est une victoire économique et culturelle décisive pour la France. Cependant, on ne peut pas vouloir rompre avec le « quoi qu’il en coûte » sans optimiser l’utilisation des deniers publics. En l’occurrence, l’essentiel est de soutenir les artisans et les PME qui recrutent et forment des apprentis, plutôt que de risquer d’entretenir une aubaine pour les grands groupes. Je ne sais pas si vous retiendrez cette mesure. J’espère en tout cas qu’elle contribuera à renforcer et à pérenniser l’apprentissage, qui est une chance pour tous nos jeunes. Je souhaite que cette disposition offre l’occasion d’une concertation avec les partenaires sociaux. occasion pour saluer M. le rapporteur général, qui a proposé plusieurs pistes pour réduire nos dépenses publiques. Notre groupe soutient cette démarche, notamment s’agissant de la maîtrise de la masse salariale de l’État. l’initiative de la commission des finances, le Sénat propose d’économiser 150 millions d’euros en réduisant les effectifs des opérateurs de l’État. Charge désormais au Gouvernement d’identifier les opérateurs qui pourront faire mieux avec moins. Il est nécessaire de réaliser ces économies, même si aucune économie n’est jamais populaire. C’est le prix à payer pour continuer à investir dans les missions régaliennes de l’État. de l’examen du projet de loi de finances, notre groupe soutient le renforcement de l’État dans ses missions régaliennes. Je me réjouis à cet égard de la hausse significative des budgets de la défense, des forces de l’ordre et de la justice. Si nous voulons rétablir l’autorité de l’État, il faut nous en donner les moyens. Alors que les menaces se multiplient, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières, ce réarmement matériel est indispensable, car c’est un préalable au réarmement moral dont nos démocraties fatiguées ont tant besoin. Réaliser des économies là où c’est possible pour investir là où c’est indispensable : telle est, mes chers collègues, la ligne que notre groupe a tenté de suivre tout au long de l’examen de ce projet de loi de finances pour 2024. C’est pourquoi, dans un esprit de responsabilité, nous avons voté la majorité des économies proposées par la commission. Toutefois, toutes les économies ne sont pas bonnes à prendre. Le rejet de plusieurs missions importantes, au premier rang desquelles les missions « Immigration, asile et intégration » et « Cohésion des territoires », ampute le budget de l’État de manière artificielle. Je regrette que la majorité sénatoriale n’ait pas fait de propositions pour adopter tous les crédits. propositions ! Ne pas adopter certaines missions, c’est ne pas assumer certains défis. Parce qu’il manque de crédits, je crains que le budget ne manque finalement de crédibilité. Cela me fait penser à une autre image qui a marqué la campagne du nouveau président argentin. On le voit passer devant un tableau où sont annotés les différents ministères de son pays. Un à un, il arrache les en criant : « », Dehors ! » C’est ainsi que les populistes s’attaquent à réduire la dette publique. Mes chers collègues, je pense qu’il existe un chemin plus raisonnable pour rétablir nos comptes. Le groupe Les Indépendants salue les économies présentées dans ce budget, mais regrette le rejet de certains crédits. C’est pourquoi, dans sa majorité,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Union Centriste est particulièrement préoccupé par l’état des finances publiques.

En matière d’enseignement, Anne Sophie Romagny a évoqué la réussite de l’apprentissage, tout en rappelant les difficultés financières de France Compétences.

du revenu des agriculteurs. Yves Bleunven a rappelé la nécessité d’une évaluation du soutien à l’investissement productif. Vincent Capo Canellas a souligné la nécessité de l’évaluation des actions du plan de relance.

Olivia Richard a regretté les délais de traitement de la justice administrative. Philippe Bonnecarrère a souligné des résultats particulièrement décevants en matière de lutte contre l’immigration irrégulière,

Nathalie Goulet a formulé de nombreuses propositions pour lutter contre l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale. Il est nécessaire d’agir plus vigoureusement en la matière, faute de quoi nous irons au devant des difficultés. Bernard Delcros vous a proposé une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus et la taxation des rachats d’actions par les grandes sociétés, qui sont très régulièrement décriés. Ce sont des propositions concrètes Sylvie Vermeillet vous a proposé de transformer l’impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « monde d’après » est désormais sous nos yeux. Nos débats n’y ont pas échappé ; ils ont clairement tourné autour de trois enjeux. Tout d’abord, nous sommes entrés dans un nouveau cycle au niveau monétaire. Il nous faut à présent anticiper des chocs d’inflation à répétition, la moindre étincelle diplomatique étant susceptible de mettre le feu aux liquidités massivement injectées depuis 2008. Avec le resserrement monétaire, les politiques budgétaires sont désormais au centre des politiques économiques. Or, de ce point de vue, un déficit de 150 milliards d’euros, soit la moitié des recettes nettes de l’État, impacte nos marges de manœuvre. Au niveau social, l’accès au logement, l’habitat et les mixités se trouvent au cœur des tensions nées de l’accentuation, d’une part, des mobilités intrafamiliales, professionnelles, migratoires et culturelles, et, d’autre part, des angoisses sociales nées du terrorisme, de la guerre, du choc des pandémies. au niveau environnemental, la planète a franchi six des neuf limites vitales, et l’effort n’est pas suffisant pour y faire face. Les accords de Paris fixaient la limite à +1,5°degré. Nous allons vers +3°degrés, et le Gouvernement nous enjoint de nous préparer à +4°degrés

Face à ces défis, que propose le Gouvernement ? Certes, il propose d’amorcer un virage pris avec la planification écologique, et c’est une première. Mais, avec seulement 7 milliards d’euros – et encore, en recyclant des crédits –, on est très loin du compte. Les inégalités sociales et patrimoniales ne font l’objet d’aucune correction : au contraire Fondamentalement, tout cela se traduit par une : « stabilité fiscale », ce qui, au passage, entretient une confusion supplémentaire – et c’est là le plus grave – entre stabilité du système fiscal et stabilité du niveau des prélèvements obligatoires. Or ni l’un ni l’autre ne résiste aux faits.

De ce point de vue, refuser d’amorcer structurellement le virage de la fiscalité écologique est coupable : coupable pour ce qui est de la planète et de la protection face aux aléas climatiques, mais coupable aussi pour ce qui est du bon état des finances publiques Qu’attendez vous, monsieur le ministre ? Pourquoi n’engagez vous pas dès maintenant un véritable virage fiscal en donnant à chacun une visibilité pluriannuelle ? Le rôle d’un État, c’est de prévoir le changement et de sécuriser ceux qui vont le vivre. De même, avoir pour objectif la stabilité du niveau de prélèvement est une erreur capitale. Il faudrait dégager près de 120 milliards d’euros supplémentaires pour être au rendez vous et du déficit, et de la transition écologique, et du service de la dette, qui va croître de 35 milliards d’euros d’ici à trois ans. ans. Dans ce contexte, vous décidez de maintenir vos objectifs de baisse des impôts, notamment de production, sans dire par quoi cette baisse va être compensée. Par l’impôt sur la consommation ?

Nous avons besoin d’un État stratège qui détermine des orientations, mobilise les moyens appropriés et fixe un cap et définisse un projet. Une politique financière ne fait pas une politique budgétaire, encore moins une politique économique, et encore moins une politique de transition écologique. De son côté, comment le Sénat a t il traité ce PLF ? Là aussi, pas de modifications structurelles : la majorité sénatoriale a fait sienne la confusion entre stabilité fiscale et stabilité du niveau des prélèvements. Elle a même voté plusieurs amendements non gagés qui enfanteront du déficit et de la dette, à l’image de la reprise du dispositif dit « Balladur » sur le logement. Faire baisser les impôts pour quelques uns par la dette pour tous est à nos yeux inacceptable. Certes, ce budget contient des avancées timides, que nous accueillons

mais non les baisser pour les baisser. De même, la fiscalité sur le patrimoine doit être revisitée, car il n’y a pas d’autre voie que de prélever les richesses qui dorment, non de manière confiscatoire, mais de manière équitable et efficace.

Enfin, dans cette période de crise, nous avons proposé de mieux soutenir le logement social. Ce modèle a fait ses preuves en 2008, au moment de la crise de la promotion immobilière,

la Banque de France prévoit un effondrement de l’investissement des ménages : –5,8 % en 2023, –5,9 % en 2024 ! L’État social continue donc de se dégrader.

Ce sont tous ces éléments qui ont conduit notre groupe à déposer une motion tendant à opposer la question préalable. Celle ci ayant été rejetée, nous avons proposé l’élaboration d’un contre budget d’initiative citoyenne constitué de plus de 150 propositions de recettes, mais aussi de relance de l’économie, des services publics et du pouvoir d’achat.

d’un même centre de gravité : des économies sur les ménages, les services publics et l’égalité territoriale, mais non sur les actionnaires ni sur les hauts revenus. Les économies se font aussi contre la planification écologique. En la matière, monsieur Cazenave, je vous cite : « Nous sommes loin de la révolution écologique. » Là dessus, soyons justes, il est impossible de douter de votre franchise… J’en viens à la dernière raison de notre vote contre : elle est motivée par l’adage classique : « Socialisation des pertes et privatisation des profits ». vous faites le choix de la dette au détriment de l’impôt. S’endetter peut être utile pour investir : c’est ce qu’on appelle une dette saine. Mais le problème est l’ampleur et la structure de la dette

part, la dette vient aussi en grande partie du refus d’une fiscalité juste et progressive pour tous. Pour la très grande majorité de nos concitoyens, le système fiscal français est progressif. Toutefois,

Voilà d’où viennent la dette et le déficit ! Avec 145 milliards d’euros de déficit et 280 milliards d’euros d’endettement, nous atteignons un record. Il faut clairement parler d’une dépendance aux marchés financiers. Cette bulle a été créée par les intérêts de la dette, qui produisent une fragilité de l’État. L’argent prend alors le dessus sur nos valeurs, ces trois valeurs qui nous lient : liberté, égalité, fraternité ! Or, je le dis, l’argent ne fait ni la Nation ni la démocratie. la dette privée des entreprises, et entre entreprises, un tabou – on n’a jamais le droit d’en parler –, représente 162 % du PIB, contre 105 % en moyenne dans la zone euro. La dette publique, à côté, fait pâle figure. Se déresponsabilisant, le Gouvernement fait le choix de la décentraliser – eh oui ! – et d’en faire supporter le poids par les collectivités et par les salariés, qui n’en sont pourtant pas responsables.

nommé la crise du logement. S’il y a bien un changement dans la politique de l’exécutif, c’est que le Gouvernement vient de s’extraire de la gestion des urgences. Le Gouvernement et la droite sénatoriale se sont finalement entendus, hier tard dans la nuit, en votant un article d’équilibre dont le solde est amélioré de 42 milliards d’euros. Tout était déjà réglé, entre pacte de fond et faux semblant de conflit.

de résistances nouvelles, populaires, larges et unitaires ; et alors, je vous le dis, tout est possible ! La parole est à M. Christian Bilhac, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Mais, contrairement au marathon olympique, dont la distance est immuable, celui là ne cesse de s’allonger, année après année, en raison du nombre croissant d’amendements déposés. Le droit d’amendement est un droit fondamental du parlementaire, sur lequel il serait dangereux de revenir. Mais peut être faudra t il encore modifier notre règlement étant donné la contrainte de durée qui encadre l’examen de la loi de finances.

Le Sénat a apporté au texte présenté par le Gouvernement de nombreuses modifications dont il faut se féliciter. Concernant la partie recettes, je tiens à souligner les avancées inscrites dans le texte par le Sénat : plus de 1,5 milliard d’euros au bénéfice des collectivités territoriales.

Je n’oublie pas l’élargissement à tout le territoire du prêt à taux zéro, qui permettra de soutenir l’accession à la propriété et le secteur du logement.

on peut s’interroger sur le sort qui, le cas échéant, serait réservé aux amendements déposés par les sénateurs en séance ou en commission. Il convient de noter que le Sénat a fait preuve de responsabilité dans l’examen de ce texte texte : si de nombreuses avancées ont été votées, en particulier en faveur des collectivités territoriales, le déficit global, lui, a été réduit par rapport au texte initial du Gouvernement. que ce déficit devient de plus en plus inquiétant, d’autant que la charge de la dette va être encore aggravée, dans les années à venir, par la hausse des taux d’intérêt.

évidence ! Au risque de me répéter, ce n’est pas sur les services publics qu’il faut s’acharner, car la population en a besoin ; c’est à notre suradministration, pléthorique et paralysante, Enfin, avec les collègues de mon groupe, je me réjouis qu’une quinzaine de nos amendements aient été adoptés. Je souligne aussi que, sur certaines missions,

La parole est à M. Didier Rambaud, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

le budget d’une majorité sénatoriale à la hauteur de ses responsabilités. À l’issue de nos soixante dix heures de débats, ce contre budget, le voilà, et il est temps de faire les comptes. Je vous assure que l’on n’est pas déçu du voyage

? Les crédits de toutes ces missions ont été rejetés, pour des raisons que je peine encore à comprendre. Vous nous dites qu’il s’agit de marquer un désaccord politique ; mais vous pouviez proposer un contre budget ! Telle était d’ailleurs votre ambition de départ, que vous n’avez cessé de répéter dans la presse.

Il n’y a plus de stratégie d’ensemble : chacun y va de son petit amendement, et des pans entiers du budget sont passés par pertes et profits pour financer les quelques dépenses consenties au profit de votre électorat. C’est cela que vous appelez un État fort, au rendez vous des défis du siècle

Mes chers collègues, cette irresponsabilité est d’autant plus regrettable que l’examen de la première partie fut l’occasion de voter des dispositions positives pour nos finances publiques.

Avances à l’audiovisuel public », sans oublier la baisse des moyens alloués à l’aide médicale de l’État, pourtant indispensable du point de vue de la sécurité sanitaire comme d’un point de vue humanitaire. Mes chers collègues, compte tenu des amendements votés en première partie et des profonds désaccords que nous avons quant aux missions rejetées en seconde partie, force est de constater que le budget qui sort du Sénat ne ressemble à rien. Il ne ressemble ni à un budget digne d’un parti de gouvernement ni même à un budget tout court ce n’est ni plus ni moins qu’un texte à trous où les failles s’accumulent ! Qu’y trouve t on ? Des politiques non financées, notamment en matière de logement ; des coups de rabot qui ressemblent plutôt à des coups de hache ; des amendements non évalués ; des économies de plusieurs milliards d’euros dont aucun contour n’est défini.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis afin de clore l’examen de ce projet de loi de finances pour 2024. Le vote que nous nous apprêtons à émettre n’a de solennel que le nom, tant, après un énième 49.3, les parlementaires que nous sommes pouvons légitimement nous interroger sur le sens de la mission pour laquelle nos électeurs nous ont élus.

Dans une société où la crise démocratique est de plus en plus prégnante, nous ne pouvons pas nous résoudre à accepter que le Parlement ne soit plus qu’une caisse d’enregistrement de décisions prises ailleurs. D’ailleurs, le cinglant camouflet que le Gouvernement a subi hier est la manifestation claire que cette méthode n’est plus acceptée, car elle est devenue trop inacceptable. Si nous ne sommes pas capables de réinventer un mode d’organisation politique qui soit plus soucieux des aspirations de nos concitoyens, alors d’autres s’en chargeront, ceux là mêmes qui laissent penser à des concitoyens crédules que le problème serait notre système démocratique. Je le dis avec force, l’effondrement des croyances associées à la démocratie représentative devrait nous préoccuper au plus haut point. Entrons maintenant dans l’analyse du texte que nous avons examiné. Je l’avais annoncé lors de la discussion générale, ce budget fait face à un triangle d’incompatibilité que trois semaines de séance n’auront pas réussi à résoudre. Durant nos débats, comme prévu, l’obsession du Gouvernement à maintenir la baisse des impôts est entrée en collision avec son obsession à réduire le déficit public. Mais, monsieur le ministre, vous n’êtes pas à une incohérence près. Ça, c’est vrai ! J’en veux pour preuve les moyens prétendument mobilisés en faveur des investissements verts, qui sont objectivement loin de répondre aux objectifs de décarbonation que vous vous êtes vous même fixés. Enfin, comme si l’incohérence n’était pas suffisance, vous avez essayé de nous convaincre que les réductions de dépenses publiques ne se feraient pas au détriment des plus fragiles d’entre nous. Mais, sur ces travées, personne n’est dupe. Pourtant, sur le papier, la promesse était alléchante. Ce budget devait être un moyen de consolider nos finances publiques tout en continuant de baisser la fiscalité et d’investir pour l’avenir. s’est une nouvelle fois fracassé sur le mur des réalités, et votre postulat de départ constitue un vœu pieux, bien éloigné du réel. Votre boussole reste la baisse systémique des impôts sur le capital. Néanmoins, je note que, pour ne pas apporter de pistes de financements nouvelles, vous avez refusé, comme chaque année depuis 2017, d’aborder des sujets structurants, comme la fiscalité du capital ou la contribution des plus aisés à l’effort collectif de redressement des comptes publics. Nous regrettons que, tout au long de nos séances, vous fussiez dans l’incapacité de sortir de votre cécité dogmatique. Que ce soit l’instauration d’un ISF vert ou la suppression de la, en passant par une réelle taxation des dividendes, rien n’aura trouvé grâce à vos yeux. Ce jusqu’au boutisme fiscal a néanmoins un coût, car votre politique de l’offre, faite de désarmement fiscal permanent, ne permet pas de réduire la dette, dont vous nous parlez tant à longueur de débat. Pour reprendre une expression chère à la majorité présidentielle, vous démontrez effectivement qu’il n’y a pas d’argent magique ; votre fragilisation de la fiscalité n’est pas tenable. À ce propos, j’aimerais vous rappeler que s’il y a bien une dette dont il faut tenir compte en priorité, c’est la dette écologique ; et celle ci n’est ni négociable, ni repoussable, ni renouvelable. raison pour laquelle nous pensons qu’au cœur du budget aurait dû figurer la bifurcation écologique. Pour atteindre l’objectif de neutralité carbone, 34 milliards d’euros sont nécessaires Les 7 milliards d’euros que vous nous avez proposés dans ce budget nous semblent bien dérisoires. Sachez que l’explication qui consiste à dire qu’ils seront multipliés dans les collectivités territoriales ou les organismes de financement public ne nous a absolument pas convaincus. Avec une mise de départ de l’État si faible,… Historique ! … comment croire à la multiplication des pains ? Cette multiplication providentielle interviendrait donc au même moment où vous demandez aux collectivités de baisser leurs dépenses. Le « en même temps » a ses limites…

Enfin, alors que l’inflation persiste et touche de plein fouet les budgets des collectivités territoriales, augmentant sensiblement leurs dépenses contraintes, vous avez refusé notre proposition d’indexation de la dotation globale La droite sénatoriale, si prompte à s’autodéfinir comme intercesseur de la défense des territoires, a brillé par son absence de soutien à notre amendement visant à donner une respiration financière à nos collectivités. Par ailleurs, l’avenir des ruralités est peu lisible tant la cacophonie qui s’est jouée durant l’examen de l’article 7 a été ridicule. De même, quand 75 % des articles du projet transmis au Sénat l’ont été sans étude d’impact, le Gouvernement porte une responsabilité forte en la matière ; une association plus appropriée des parlementaires aurait permis d’éviter cet écueil. Monsieur le ministre, tout cela fleure bon l’amateurisme. Sur plusieurs sujets majeurs, au final, personne n’y a rien compris. Je souhaite que l’atterrissage sur les zonages des ruralités, comme sur d’autres questions, se fasse le plus en douceur possible en intégrant les demandes légitimes des territoires. Il est un autre atterrissage dont l’issue me semble incertaine : c’est celui du devenir de nos amendements votés sur ces travées après de nombreuses heures de séance. Cela me permet de revenir à mon point de départ : quelle démocratie voulons nous en France en 2023 ? Pour ne prendre que quelques exemples concrets, monsieur le ministre, allez vous balayer d’un revers de main notre amendement visant à prévoir 350 millions d’euros supplémentaires en faveur des mesures agroenvironnementales et climatiques ? Allez vous revenir sur la suppression de cette scandaleuse niche fiscale pour la Fifa, instaurée à l’Assemblée nationale ? Allez vous maintenir le PTZ pour les primo accédants sur l’ensemble des territoires, comme nous vous l’avons proposé ? Allez vous accepter le maintien du fonds de soutien aux activités périscolaires, que nous jugeons très important ? Autant d’exemples sur lesquels la balle est dans le camp du Gouvernement, monsieur le ministre. Parce que nous ne nous faisons aucune illusion, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera contre ce budget, tant il nous apparaît inique, à sens unique et incapable de nous permettre de relever la complexité des problèmes contemporains s’imposant à nous.

au sort la lettre par laquelle commencera l’appel nominal.

040 amendements l’an dernier. Malgré les évolutions engagées depuis deux ans, force est de constater qu’il devient de plus en plus difficile d’assurer la qualité de nos débats

Pour l’heure, je souhaite remercier tout particulièrement le rapporteur général de la commission des finances, Jean François Husson, de son écoute et de la qualité de son travail ; ses avis ont permis à chacun de se prononcer en pleine connaissance de cause.

Il a contribué par sa particulière vigilance et sa pédagogie à ce que les temps d’examens soient respectés, ce qui n’était pas gagné au départ. Je veux également remercier les présidentes et les présidents de séance, qui ont permis que nos débats se déroulent de manière apaisée. Je salue les 49 rapporteurs spéciaux de la commission des finances, les 76 rapporteurs pour avis des autres commissions, ainsi que les présidents de ces dernières et les chefs de file des huit groupes politiques, pour leur contribution à nos débats. Je remercie

confirmer que notre démocratie est aujourd’hui fragile. Nous devons plutôt, comme nous le faisons au Sénat depuis un certain temps, faire en sorte qu’elle puisse vivre en nous écoutant les

de l’éducation et de la communication, l’examen de la proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat afin de compléter l’intitulé de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, présentée par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues Dans la discussion générale, la parole est à M. Laurent Lafon, auteur de la proposition de résolution. Monsieur

je me réjouis que la conférence des présidents ait accepté d’inscrire à l’ordre du jour de notre assemblée l’examen de cette proposition de résolution visant à compléter l’intitulé de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, que j’ai l’honneur de présider depuis le mois pour y ajouter le mot : « sport ». C’est une modification que certains d’entre nous appelaient de leurs vœux depuis plusieurs années. Grâce au soutien résolu du président du Sénat, elle est sur le point de se concrétiser.

Dans l’esprit de mes trois collègues, comme dans celui de l’ensemble de ses signataires, cette proposition de résolution ne se limite pas à l’adoption d’une simple variation sémantique autour des compétences de la commission de la culture. La modification du règlement du Sénat qui vous est proposée aujourd’hui vise aussi et, surtout, à souligner la place que notre assemblée accorde désormais au sport dans ses travaux. Au cours de ces vingt dernières années, effet constaté que le sport est devenu une matière législative à part entière, et ce n’est ni le président de la commission des lois, qui a souhaité – et obtenu – de pouvoir examiner au fond le dernier projet de loi sur les jeux Olympiques et Paralympiques ni celui de la commission des affaires sociales, chargé d’examiner chaque année des amendements au projet (PLFSS) visant à la prise en charge du « sport santé », qui me contrediront. Le rapport réalisé par François Noël Buffet sur cette proposition de résolution rappelle, de manière opportune, que, depuis le début des années 2000, pas moins de vingt quatre textes consacrés au sport ont été examinés au fond ou pour avis par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, représentant près de 10 % de son activité législative annuelle. Cette hausse du nombre de textes examinés chaque armée par la commission et le Sénat illustre la place grandissante prise par le sport, son organisation, sa promotion, son économie, voire ses dérives, dans la vie de notre pays, de nos collectivités et, bien évidemment, dans celle de nos concitoyens. La matière est riche et reflète les préoccupations de notre temps. Les textes qui en relèvent traitent aussi bien du sport amateur que du sport professionnel, visent à réglementer le statut juridique des arbitres comme celui des agents des joueurs, entendent lutter contre le trafic de produits dopants et promouvoir l’éthique et les droits des sportifs, tendent à réprimer le hooliganisme et à garantir la protection des mineurs et de l’honorabilité des encadrants bénévoles. Si l’activité législative de la commission – et du Sénat – consacrée aux thématiques du sport s’est accrue, il en va de même en matière de contrôle. La commission a ainsi lancé, au cours des dernières années, des travaux traitant à la fois de problématiques transversales, comme celle des politiques territoriales du sport, de questions spécifiques, comme la situation des conseillers techniques sportifs, mais aussi de questions d’actualité, à l’image de la mission commune d’information, menée conjointement avec la commission des lois, consacrée aux incidents survenus en marge de l’organisation de la finale de la Ligue des champions de football au Stade de France le 28 mai 2022.

la commission s’est, comme d’autres, saisie de la question des jeux Olympiques et Paralympiques, en lien étroit avec la Cour des comptes, afin d’en contrôler les modalités d’organisation, mais aussi d’en comprendre les conséquences sur d’autres pans de ses compétences en particulier à l’organisation des événements culturels, notamment des festivals, au printemps et à l’été 2024. Au regard de la place prise par le sport au sein de l’activité législative et de contrôle de la commission et, plus largement, au sein de notre institution, et au moment où notre où notre pays s’apprête à accueillir le principal événement sportif de la planète, j’espère, mes chers collègues, que le Sénat adoptera à l’unanimité cette proposition de réforme de son règlement. La parole

qu’elle a adoptée sans modification. Cette proposition de résolution a pour objet de modifier les dispositions de l’article 7 du règlement du Sénat, qui traite du nombre, de l’intitulé et des effectifs des commissions permanentes, afin de mentionner le sport dans l’intitulé de la commission que préside notre collègue Laurent Lafon. Celle ci deviendrait alors la commission « de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport

avant que son intitulé ne trouve sa formulation actuelle à l’occasion de la réforme du règlement du Sénat du 2 juin 2009. La volonté du Sénat, en 2009, d’octroyer un intitulé plus complet à l’ancienne commission des affaires culturelles s’est justifiée par le choix fait dès fait dès 1959 de ne pas préciser, au sein du règlement du Sénat, les compétences des différentes commissions permanentes, contrairement à la pratique de l’Assemblée nationale. Ce choix, gage d’une certaine souplesse et d’un dialogue constant entre commissions, confère cependant une importance d’autant plus grande aux dénominations des commissions, qui doivent exprimer leurs attributions sans excès d’exhaustivité, mais de façon claire et englobante. C’est dans cet état d’esprit a déterminé sa position sur cette proposition de résolution. Or nous constatons que le sport constitue une compétence traditionnelle de la commission de la culture,

la commission a publié dix rapports d’information sur des sujets liés au sport, ce qui représente 7,2 % des rapports d’information publiés sur cette période. Nous avons donc considéré que la proposition de modification du règlement qui nous réunit aujourd’hui est cohérente au regard de la part du sport au sein de l’activité législative et de contrôle de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication ; c’est probablement l’une des dernières fois qu’on l’appellera ainsi. Cette nouvelle dénomination participerait, en outre, à moins de huit mois du lancement des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, à accorder davantage de visibilité au sport dans les travaux de notre institution et à démontrer l’attachement que porte le Sénat à la bonne tenue et à la réussite de ces jeux.

Enfin, nous avons pris note du caractère très largement transpartisan de cette proposition de résolution, puisqu’elle a été cosignée par quarante quatre collègues membres de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication – c’est la dernière fois que je prononce son intitulé de façon incomplète –, issus de l’ensemble des groupes politiques représentés au Sénat. Pour toutes ces raisons,

Le Sénat n’a pas attendu la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour s’intéresser de près au sport : c’est dans le temps long que la chambre haute a progressivement marqué son attention et son attachement aux politiques publiques sportives et au développement de la pratique en France, son rôle législatif. pour ne parler que de ces dernières années, nous avons débattu et adopté plusieurs lois pour accompagner la préparation des jeux de 2024, pour démocratiser le sport en France, en posant les jalons d’une meilleure pratique quotidienne d’une activité physique ou sportive et en accompagnant les fédérations sportives dans l’évolution de leur gouvernance, pour assurer une meilleure représentativité de leurs instances internes. Le Sénat a également voté des progrès sur des textes à portée plus générale. Je pense d’abord à la réforme des retraites, par laquelle nous avons élargi le dispositif de rachat de trimestres pour les retraités sportifs de haut niveau.

les collectivités nous font part chaque jour de leurs difficultés pour assurer leurs missions de service public sur le financement des équipements structurants ! De nombreux événements ont aussi animé la vie du Sénat, à l’instar de la présentation du dispositif Terre de Jeux pour les jeux Olympiques et Paralympiques et des 100 ans du maillot jaune. La Haute Assemblée a aussi accueilli les médaillés des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver et d’été, et organisé la journée olympique, en juin dernier, pour présenter les nouvelles disciplines dans le jardin du Luxembourg.

la part budgétaire de l’État consacrée à ces politiques, qui représente aujourd’hui moins de 0,2 % des crédits, il nous faut travailler pour relever le plafond des taxes affectées provenant des paris sportifs et autres ressources issues du sport, mais aussi sur une harmonisation des taux de TVA de l’économie du sport et, enfin, sur une évolution et un meilleur accompagnement du financement privé de la pratique sportive. Dans notre mission de contrôle, nous devons être vigilants à l’application des mesures adoptées par le Parlement s’agissant de la gouvernance des fédérations, mais aussi des sujets d’actualité, comme l’éthique, la parité et les violences dans et autour du sport. Il nous faut également répondre aux difficultés des collectivités. Nous pensons ainsi qu’il faudrait mettre en place un véritable plan Marshall, en partenariat avec les régions, départements et autres collectivités locales, ce qui est des équipements structurants, notamment les piscines, comme cela avait été engagé dans les années 1970. Notre pays accueille les jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 et va organiser ceux de 2030 dans les Alpes. Profitons de ces deux événements planétaires pour promouvoir et assurer une pratique régulière de tous, développer le sport à l’école, impulser la pratique d’activités physiques en direction du monde de l’entreprise, soutenir les associations et les millions de pratiquants et de bénévoles, déployer le sport santé, avec la prise en charge de l’activité physique adaptée pour certaines maladies. Surtout, dans le cadre de ces deux événements, ne ratons pas la marche de l’héritage, sous peine d’attendre à nouveau des décennies pour donner au sport la place qui devrait être la sienne dans les politiques nationales. La Chambre haute a eu à cœur d’œuvrer à une plus grande pédagogie et à une promotion de la pratique sportive. En dehors des moments législatifs et des événements, le Sénat est la seule assemblée à avoir un groupe d’études consacré aux pratiques sportives et aux grands événements sportifs. C’est désormais la première chambre du Parlement à offrir au sport une vraie reconnaissance au travers du nom de l’une Je tiens à remercier le président de celle ci, Laurent Lafon, de son soutien, son écoute et son engagement sur tous les sujets qui concernent le sport. Enfin, je veux souligner le soutien sans faille et le suivi du président Larcher sur tous les enjeux qui touchent à la pratique sportive et aux grands événements qui se déroulent sur nos territoires.

mes chers collègues, nous avons, au Sénat, la volonté de faire de notre pays une « nation sportive ». Aussi, au vu de l’importance croissante que prend le sport dans nos travaux parlementaires et dans la vie du Palais du Luxembourg, il était logique de signifier symboliquement toute la place qu’il prend désormais, en l’intégrant pleinement dans l’intitulé de notre commission.

Le contexte – il faut le bien le reconnaître – est particulièrement favorable. Après avoir reçu les passionnés de rugby du monde entier lors de la Coupe du monde, notre pays s’apprête à accueillir à Paris les prochains jeux Olympiques et Paralympiques. La France pourrait également organiser les jeux Olympiques d’hiver 2030 si la candidature des Alpes françaises était définitivement ratifiée par le Comité international olympique, au mois de juillet 2024. L’un comme l’autre sont des événements d’envergure mondiale, présentant des défis multiples. Ils nous invitent à nous projeter dans l’avenir et à œuvrer collectivement pour faire de la France une grande nation sportive. Pour donner corps à cette ambition, nous savons que nous pouvons compter sur la mobilisation des élus locaux et de l’ensemble du réseau associatif, éducatif et médical. À cet égard, je tiens à rendre hommage aux nombreux bénévoles qui s’investissent dans nos villes et nos villages, pour transmettre les valeurs et la passion du sport. À leurs côtés, nous serons mobilisés pour faire vivre l’héritage des jeux, bien au delà de la cérémonie de clôture. Dans la perspective de l’année historique à venir, et pour un avenir désirable, nous devons généraliser la pratique du sport dans tous les territoires. Il s’agit d’un facteur essentiel de cohésion nationale, mais aussi d’un enjeu de santé publique. À cet égard, je veux saluer le nouveau plan « 5 000 terrains de sport – Génération 2024 », qui bénéficiera aux équipements sportifs de proximité et aux cours d’école. Ce plan, qui prolonge un premier plan ayant permis de rénover et de créer 5 000 plateaux multisports, aires de fitness et terrains de basket, permettra de concrétiser l’ambition de promotion de l’activité physique et sportive dès le plus jeune âge. Il accompagne idéalement la mesure mise en place pour la pratique d’une activité physique quotidienne de trente minutes à l’école. La passerelle entre sport et éducation et entre sport et santé est indéniable : il n’est pas permis d’envisager l’un sans les autres. La commission se mobilise depuis longtemps, avec une constance et une conviction jamais prises en défaut, en faveur du sport pour tous, à tous les âges de la vie. Au Sénat, le champ de compétences de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication dépasse donc largement son seul énoncé. Les enjeux du sport et de ses acteurs faisant partie de nos sujets de travail majeurs, le nom de la commission doit refléter pleinement cette réalité. Pour cette raison, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de la présente proposition de résolution, visant à compléter l’intitulé de la commission. La parole

Monsieur le président, mes chers collègues,

vise à adjoindre le sport à l’intitulé de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, en modifiant l’article 7 du règlement du Sénat. Loin de constituer une démarche exceptionnelle, le présent texte reflète l’évolution de l’environnement dans lequel opèrent les commissions. et de faire correspondre leur intitulé à la réalité de leurs travaux, tant législatifs que de contrôle, comme ce fut le cas en son temps, pour cette même commission, avec la réforme du règlement du 2 juin 2009. D’aucuns pourraient soulever le peu de substance, voire la vacuité, de cette démarche au regard des travaux concrets de la commission. Effectivement, on peut considérer que tout est dans tout, et réciproquement mais cela va mieux en le précisant ! Je ne vous apprendrai pas, mes chers collègues, l’importance du poids des mots, surtout quand ils ne laissent que peu de place à l’interprétation, entérinant certes une situation de fait, mais avant tout une compétence traditionnelle de la commission. Cette approche nous oblige en tant que législateurs, et c’est le sens de cette proposition de résolution. Au delà, il s’agit surtout d’acter un constat : l’importance du sport aujourd’hui. Certes, à moins de huit mois du coup d’envoi des prochains jeux Olympiques et Paralympiques, cette modification revêt avant tout une dimension éminemment symbolique. Mais elle traduit également, me semble t il, l’envergure du sujet, à la fois, pour les acteurs du monde sportifs, pour nos territoires et pour notre société. Ne pas l’affirmer aurait constitué un manquement, surtout à l’heure où le Président de la République prône le sport comme grande cause nationale en 2024. Pour ma part, particulièrement investi depuis des années sur les questions relatives au sport dans toute sa diversité et toutes ses problématiques, je m’inscris totalement dans cette démarche. Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, j’invite l’ensemble de mes collègues à faire de même.

Monsieur le président, Monsieur le président, mes chers collègues, nous examinons ce jour une proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat, afin de compléter l’intitulé de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Le sport occupe aujourd’hui une place importante dans le cœur des Françaises et des Français. Ciment de notre société, il est un bien précieux d’émancipation, de socialisation et de solidarité. Sa place croissante reflète les attentes de nos concitoyennes et concitoyens sur le sujet, des attentes visibles au travers de nos débats au Sénat. L’histoire de notre institution montre quelle place significative est consacrée au sport dans l’activité constante de notre commission.

un symbole fort pour nos collectivités territoriales, qui sont au cœur des pratiques en termes d’équipements, d’encadrement et de soutien aux clubs. Elles sont en effet, au quotidien, les interlocutrices du monde sportif et mènent avec lui des missions d’intérêt général autour de la pratique physique. Inscrire le sport dans l’intitulé de notre commission sénatoriale serait aussi rendre hommage à l’ensemble des élus qui agissent sur le terrain. Ce serait un symbole fort, aussi, pour rappeler l’importance de la pratique physique au quotidien. Le sport ne doit pas être envisagé comme un sujet de niche.

Les écologistes considèrent que le sport est un enjeu global, qui doit être perçu et appréhendé en lien avec les attentes de notre société. Il s’agit d’une lutte de chaque instant pour sortir les jeunes de la sédentarité, pour développer la tolérance, pour pérenniser le cadre populaire des activités sportives et pour lutter, encore et toujours, contre les violences sexistes et sexuelles. Le sport est également une vitrine de nos combats politiques. Quelle place lui faisons nous dans un monde qui se dirige vers un réchauffement de plus de 2,5 degrés à la fin du siècle ? Il est urgent de penser le sport de demain. Notre rôle, en tant que parlementaires, est d’être force de proposition pour garantir une pratique sportive durable et soutenir à chaque instant nos collectivités dans cette transition.

Monsieur le président, mes chers collègues, en cette pré année olympique, alors que Paris s’apprête à devenir la capitale de tous les athlètes du monde, il était paradoxal que notre Haute Assemblée n’affiche pas, dans la dénomination

tous les milieux sociaux. Plus encore, il participe à la diffusion des principes essentiels au bon fonctionnement de la République, et plus globalement de la société. Bien évidemment, je placerai en tête de ces principes le respect des partenaires et des adversaires, ainsi que le dépassement de soi au bénéfice du collectif. La pratique sportive demeure un espace de mixité sociale et culturelle qu’il convient de consolider et de renforcer, d’autant plus dans la période actuelle, où le repli identitaire et le refus de l’altérité progressent dans de trop nombreux pans de la société. En effet, sous les mêmes couleurs et les mêmes maillots, chacune et chacun dispose des mêmes chances de s’épanouir, d’exprimer l’ensemble de ses capacités et de se sentir membre d’un collectif. Ce travail de fond si essentiel, infusé dans la quasi totalité de la population dès le plus jeune âge, est porté par des centaines de milliers de bénévoles, des milliers de clubs et d’associations et des centaines de fédérations.

Pour de nombreux jeunes enfants, le sport à l’école est non seulement un cadre d’apprentissage, mais aussi un espace de liberté et d’affirmation, dans lequel les déterminismes sociaux et familiaux s’atténuent.

contraire, d’une activité constitutive de la condition humaine, depuis que nos ancêtres préhistoriques ont couru, sauté, lancé, grimpé et se sont affrontés non seulement pour se nourrir ou survivre, mais aussi pour s’entraîner à être plus performants dans leurs activités de chasse et de survie,

mais qui sont des épreuves individuelles ou collectives contre le temps ou des adversaires. Après l’exhibition des vertus de la noblesse ou l’affrontement grégaire de rivalités villageoises, l’époque victorienne et réglementer le sport pour sélectionner les futurs leaders appelés à dominer le monde, plutôt que de s’en remettre aux seules élites universitaires. le sport a été rattrapé par la fièvre économique, du fait de la professionnalisation de certaines disciplines et de leur marchandisation. Il ne peut plus être géré par la seule sphère privée

tout naturellement de reconnaître la place du sport en ajoutant ce noble mot à l’intitulé de notre commission.

c’est une proposition de résolution pleine de bon sens que nous examinons. Je ne suis sans doute pas le seul, en effet, à m’étonner que le sport soit encore exclu de l’intitulé de la commission du Sénat dédiée à la culture, à l’éducation et à la communication.

consacrés au sport, dont trois relatifs à l’organisation des prochains jeux Olympiques et Paralympiques ? Pourquoi ne pas modifier le règlement du Sénat, alors même que cette commission a pris l’initiative de lancer cinq missions de contrôle, sur le thème du sport, sur les politiques territoriales du sport ou encore sur la situation des conseillers techniques sportifs ?

l’inclusion. « Le sport, parce qu’il gomme les inégalités, est un catalyseur de la cohésion sociale »,

Ce volontarisme, accompagné de celui du président du Sénat et du président de la commission de la loi, a porté ses fruits. Les chiffres parlent d’eux mêmes. Avec 15,6 millions de licenciés, un chiffre encore plus élevé de pratiquants libres, 360 000 clubs associatifs, 3,5 millions de bénévoles, 119 fédérations agréées par le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et un poids économique de 71 milliards d’euros, soit 2,6 % du PIB – autant que le secteur de l’hôtellerie restauration le sport est le premier mouvement social de France. Il a toute sa place dans l’intitulé d’une commission permanente du Sénat. À cet égard, notre commission de la culture s’est régulièrement préoccupée des véritables enjeux d’une politique nationale du sport, dont la place reste insuffisante dans le débat public et politique du pays. Le match qui oppose le sport à ses dérives, parmi lesquelles le dopage, passera inévitablement par une redéfinition des liens entre le sport et l’argent, sujet ô combien tabou. Sur le plan géopolitique, de nouveaux pays déploient un particulièrement agressif : le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis prennent le relais de la Russie et de la Chine. internationaux (Gési), notamment, ne saurait relâcher ses efforts ; elle doit rester fidèle à une histoire, celle de la création par un Français des trois plus grands événements sportifs internationaux : les jeux Olympiques, la Coupe du monde de football, le Tour de France cycliste. Sur la scène internationale du sport, le maintien de l’excellence française est essentiel. Le Parlement ne peut rester à l’écart de tous ces enjeux, d’où l’importance de notre débat de ce jour. Le sport est en effet un apprentissage des valeurs collectives, mais également un formidable vecteur de messages. La présence massive du sport comme fait social est un révélateur des mutations de notre société mondialisation, financiarisation, gigantisme, métropolisation, société de l’image et du divertissement, violences, individualisme… Dans

Le risque de confusion est sans doute réel, mais la lisibilité nous impose la simplicité. La prise en compte du sport dans la vie de la Nation résulte d’une vision, celle de la place du corps dans la société. Cette problématique devient enfin d’actualité avec l’intérêt porté à la démarche Sport, santé, bien être et à son triptyque : la santé physique – être bien dans son corps –, la santé mentale – être bien dans sa tête –, la santé sociale – être bien avec les autres. Malheureusement, cette appréhension unitaire de l’homme fut longtemps entravée par une conception philosophique prédominante jusqu’au XX siècle, celle de Descartes et de son dualisme : le corps d’un côté, l’esprit ou l’âme de l’autre. Aujourd’hui, de nombreux chantiers restent ouverts, parmi lesquels la faiblesse budgétaire, l’insuffisance du nombre d’heures d’EPS dans notre système éducatif ou la réduction des inégalités sociales et territoriales d’accès à la pratique, qu’elle soit fédérée ou libre.

je regrette que le secteur de la vie associative ne soit pas intégré dans l’intitulé de notre commission. En effet, ce secteur occupe 13 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés, au sein de près de 1,5 million d’associations

médicale et caritative, etc. Cette activité associative, parallèle au système économique, constitue souvent le fondement de la vie sociale locale et permet de rassembler des personnes parfois isolées,

Mes chers collègues, en accord avec les commissions concernées et le Gouvernement, nous pourrions, demain, si l’espace réservé au groupe Écologiste – Solidarité et Territoires se terminait avant trente, tenir le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2023 avant vingt deux heures. Par ailleurs, concernant l’ordre du jour jeudi 14 décembre, nous pourrions commencer l’espace réservé au groupe Union Centriste dès la fin de celui qui est réservé au groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, si celui ci se terminait avant seize heures. Y a t il des observations ?…

Merci,